sur la santé économique des entreprises et des effets collatéraux sur l'emploi.

et des précédents projets de loi de finances. Si jusqu'à présent nos votes n'ont pas été suivis d'effet du côté du Gouvernement, nous pouvons peut-être espérer que cela change ... Non ! Depuis l'adoption de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les collectivités disposent de compétences clés et participent de façon décisive à la lutte contre le changement climatique, grâce aux plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), à l'échelle intercommunale, et aux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet),

5 euros par habitant. Cette affectation viendrait en complément de l'enveloppe de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL). Une partie serait consacrée à la transition écologique et devrait être décaissée en 2022 au titre du plan de relance,

C'est au niveau des territoires que l'on peut contribuer à la transition écologique. Mais les collectivités se sont vu transférer de nouvelles compétences sans aucun nouveau

comporter l'effet pervers de récompenser avec les ressources de l'État les collectivités n'ayant pas mobilisé leurs propres bases en instituant un versement mobilité. D'une certaine manière, aucune collectivité n'aurait intérêt à instituer le versement mobilité, ce qui reviendrait à faire supporter par l'État seul une part croissante du financement des autorités organisatrices des mobilités.

proposons de créer une réfaction de la TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l'objectif de réduction du stockage fixé par le Gouvernement, c'est-à-dire qui ont divisé par deux la masse des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010.

accompagne les collectivités pour réduire les déchets résiduels. Cette mesure, travaillée avec l'association Amorce, permettrait de répondre à l'objectif affiché par l'État de développer l'économie circulaire, plutôt qu'à simplement lui apporter de nouvelles recettes au détriment des collectivités. Quel est l'avis de la commission

de la majorité sénatoriale et ceux du Gouvernement ! Cette collusion est simple : on ne touche pas aux bénéfices des fournisseurs et on neutralise le gel des tarifs du gaz en prévoyant des mesures de compensation pour ces mêmes fournisseurs.

La mise en place de critères de moralité financière est indispensable à la lutte contre la fraude- un engagement également important.

a été transposée en droit français, dans le code général des impôts, mais elle n'a pas encore été appliquée en raison d'un délai accordé par la direction de la législation fiscale. Ce nouveau régime de TVA va poser des difficultés aux salles de cinéma, en les contraignant à refacturer la TVA aux émetteurs des contremarques qu'ils acceptent. l'exploitant devra vérifier s'il s'agit ou non d'un bon à usage unique. Le régime de TVA existant est fiable et constitue un formidable outil de promotion du cinéma dans l'ensemble du territoire. D'où l'idée d'assimiler les bons à usage unique aux bons à usage multiple, afin de permettre aux cinémas de ne pas

Il prévoit notamment de distinguer deux cas de figure : l'alinéa a, qui précise qu'en cas de versement préalable d'un acompte la taxe devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé, et l'alinéa b, qui ne prévoit pas de telles précisions. L'exigibilité de la TVA au moment de l'acompte induirait une forte pression sur la trésorerie de nombreux commerces d'équipements ménagers, ce qui semble malvenu en période de reprise économique. C'est pourquoi cet amendement vise à supprimer la distinction entre ces deux cas de figure, en ne retenant que

Cette discrimination, que la France est seule à pratiquer, j'y insiste, est totalement injustifiée et anormale d'un point de vue tant économique que nutritionnel.

L'article 9 du projet de loi de finances pour 2022 vise notamment à simplifier la lisibilité des règles fiscales en matière de TVA pour les produits destinés à l'alimentation humaine. Cet amendement est en

par cet amendement de supprimer la distinction fiscale introduite à l'article 298 du CGI et de maintenir un taux réduit de TVA pour toutes les boissons ayant les mêmes titres alcoométriques inférieurs ou égaux à 1,2

crête. Un rescrit fiscal ancien fixe à 3 kilowatts crête le seuil d'assujettissement à la TVA à taux plein pour les projets solaires. Pour tenir compte des évolutions de puissances des modules solaires, nous proposons d'adapter dans la loi la doctrine administrative aux réalités du marché. En effet, la puissance des installations solaires résidentielles se situe maintenant entre 0 et 9 crête. Le seuil existant ne correspond plus aux réalités du marché, et entraîne une limitation des capacités installées, en poussant les autoconsommateurs à sous-dimensionner leurs installations.

les normes européennes ne permettent pas de sortir des opérations économiques de la base d'imposition de la TVA. Par ailleurs, si nous devons encourager le développement de l'autoconsommation, il nous faut aussi prendre garde

à 10 %, au lieu de 20 %. Il s'agit d'un exemple concret qui permettrait de conjuguer l'exigence sociale et écologique, en rendant financièrement accessible ce qui est écologiquement responsable. Quel

Cet amendement vise à exonérer de TVA les prestations de remplacement pour congés maternité, paternité ou adoption des agriculteurs. Lors d'une naissance ou d'une adoption, les paysans bénéficient d'une allocation de remplacement permettant de financer la mise à disposition d'un salarié pour effectuer les travaux sur leur ferme durant toute la durée du congé. Le mécanisme actuel permettant l'accès à ce dispositif

outre, instaurer une exonération pour les prestations de remplacement pénaliserait les prestataires qui ne pourraient plus déduire l'intégralité de la taxe sur leurs achats. Ces mêmes employeurs seraient aussi susceptibles d'être redevables de la taxe sur les salaires frappant les personnes qui effectuent des activités non soumises à la TVA. Ce jeu de contradictions conduit le

Cet amendement vise à faire passer le taux de TVA applicable à l'ensemble des transports publics collectifs de voyageurs du quotidien de 10 % à 5,5

afin de faire diminuer les coûts et d'inciter le consommateur à utiliser ce service. Il s'agit de favoriser l'allongement de la durée de vie des produits, qui doit être l'un de nos objectifs majeurs en termes de transition écologique et économique. Quel est l'avis de la commission

aux couches pour nourrissons un taux réduit de TVA à 5,5 %, au lieu de 20 % actuellement. L'accès à des produits d'hygiène pour les nourrissons à un prix abordable est un enjeu lié à la santé des nourrissons : il s'agit d'éviter des risques d'infection Les nourrissons peuvent entrer dans la catégorie des incontinents, catégorie à laquelle la Commission européenne reconnaît un droit d'accès au taux de 5,5 % pour les protections absorbantes. L'enjeu de santé publique est indéniable et cette mesure représente aussi un soutien à la politique familiale.

celui-ci entraînant inexorablement une hausse du nombre de personnes souffrant d'incontinence urinaire. Il s'agit ici de réduire une charge financière incompressible pour le bien-vivre de nos aînés, mais aussi de certaines personnes en situation de handicap. Pour nombre de nos concitoyens, ces solutions palliatives absorbantes sont des produits de première nécessité, non de confort. Elles représentent un poste de dépenses très élevé, que certaines aides ne permettent pas de couvrir. Le coût d'achat de ces protections peut grimper jusqu'à 300 euros par mois pour les incontinences lourdes, selon l'Institut national de la consommation. Faute d'argent, des malades et personnes en situation de handicap renoncent à les acheter, même si elles sont indispensables à leur hygiène et leur bien-être. Cette proposition n'est pas contraire au droit de l'Union européenne, car les États membres peuvent appliquer un taux réduit de TVA aux produits pharmaceutiques et à certains dispositifs médicaux que sont les produits contre l'incontinence. D'ailleurs, la Belgique et les Pays-Bas appliquent déjà un taux de TVA réduit sur les protections palliatives absorbantes.

aux produits issus du commerce équitable, défini par la loi de 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, un taux réduit de TVA afin de rendre plus accessibles aux consommateurs des produits de qualité, socialement et écologiquement responsables. Il s'agit aussi par cet amendement de soutenir et de valoriser les entreprises à impact social et environnemental positif que représente le secteur du commerce équitable. En effet, en plus de garantir une rémunération juste aux producteurs, le commerce équitable accélère les investissements dans l'agriculture biologique et l'agroécologie. La fiscalité doit être un levier de transition agroécologique : la modulation du taux de TVA est dans ce cadre un levier à saisir.

la musique, le cinéma ou encore le jeu vidéo restent soumis au taux normal de 20 %. Quel est l'avis de la commission

quant à la taxation discriminante de produits de gastronomie française considérés de luxe. Pourquoi le caviar serait-il aujourd'hui le seul produit alimentaire de luxe à se voir Si ce taux pouvait se justifier à l'époque où l'on importait le caviar, ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'il est produit dans notre pays.

En effet, les produits issus de l'agriculture biologique contribuent positivement à la qualité de l'eau, des sols, de l'air et des aliments, à la protection de l'environnement, à la santé, au bien-être animal, à l'emploi et au revenu agricole. Ainsi, ces produits sont générateurs d'externalités positives pour l'environnement, la biodiversité et les territoires. Il convient donc d'en assurer la plus grande accessibilité pour tous et d'encourager leur consommation. et la fin du financement national de l'aide au maintien sont venues limiter fortement les soutiens publics à ce secteur, il nous faut, au contraire, réorienter notre politique fiscale vers l'appui à ce mode de production essentiel pour notre souveraineté alimentaire et notre transition agroécologique. L'adoption de cet amendement permettrait également de contribuer efficacement aux objectifs du Pacte vert européen, à savoir 25 % de surfaces en agriculture biologique d'ici à 2030.

En effet, ils permettent aux producteurs de fixer un prix à la fois rémunérateur pour eux et accessible au consommateur, la limitation des intermédiaires. En cultivant le lien entre consommateurs et producteurs, les circuits courts permettent également de développer des systèmes de production plus vertueux en termes de respect de l'environnement et du bien-être animal. Ils permettent aussi de relocaliser notre consommation, alors que nous importons une part

janvier 1991, accordaient des taux réduits inférieurs à 5 % pour des raisons d'intérêt social bien définies et en faveur des consommateurs finaux peuvent continuer à les appliquer. C'est le cas en France du taux dit super réduit

La vie chère constitue un élément de rupture d'égalité entre les citoyens d'outre-mer et ceux de la France hexagonale. Je parle bien de rupture d'égalité

aux tenues de protection adaptées à la lutte contre la propagation du virus et au gel hydroalcoolique. La commission des finances, sous l'autorité de son président et de son rapporteur général,

; d'autre part, lorsque les travaux d'amélioration à réaliser sur l'immeuble ancien en vue de sa transformation en logements sociaux sont effectués, non pas par l'organisme acquéreur, mais par le vendeur dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover. L'amendement n° I-28, présenté

Ces opérations permettent la création de nouveaux logements sociaux à partir de la transformation d'immeubles anciens de bureaux ou de logements privés. L'article 9 du PLF pour 2022, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit d'élargir ce régime aux opérations d'acquisition-amélioration financées par Cet amendement, déposé en lien avec l'Union sociale pour l'habitat (USH), vise à rendre cette nouvelle mesure plus opérationnelle, en prévoyant qu'elle s'applique également lorsque les travaux d'amélioration à réaliser sur l'immeuble ancien en vue de sa transformation en logements sociaux sont effectués, non pas par l'organisme acquéreur, mais par le vendeur dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover. Cette situation se rencontre régulièrement, notamment dans les zones tendues, où les montages réalisés sur des immeubles anciens sont souvent complexes.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

Cet amendement est largement compatible non seulement avec les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, mais également avec le rapport du Haut Conseil pour le climat, qui fait de l'habitat un enjeu majeur de transition écologique. Je souligne qu'un tel taux réduit a déjà été appliqué de 1999 à 2012. Il a été apprécié tant par les professionnels de la construction que par les particuliers. Aujourd'hui, seuls les travaux de rénovation énergétique sont éligibles à ce taux réduit.

qui répondent aux besoins de nos concitoyens. À cet effet, cet amendement vise à rétablir le taux de TVA de 5,5 % pour l'ensemble des opérations de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux financés par des PLAI et des PLUS, quel que soit leur lieu d'implantation.

La loi de finances pour 2018 a porté de 5,5 % à 10 % le taux de TVA pour les logements locatifs sociaux neufs. Puis, après accord avec les organismes du secteur, la loi de finances pour 2020 a abaissé à 5,5

Ils reviennent donc sur l'accord que je viens de mentionner. Il me paraît plus pertinent de favoriser les opérations les plus sociales par un taux de TVA plus bas, alors que ces amendements mettent sur un même plan les logements sociaux destinés à des

a pour objet de faciliter les initiatives de construction de nouveaux établissements de santé, notamment les centres de soins de suite et de réadaptation, en appliquant à la livraison à soi-même des constructions

à 5,5 % pour l'ensemble des travaux de rénovation énergétique réalisés dans les logements sociaux existants. Cette mesure a pour objectif de soutenir l'effort des bailleurs sociaux pour accroître la performance énergétique de leur patrimoine, permettant ainsi une baisse des charges supportées par les locataires du parc social.

seule une liste restreinte de travaux de rénovation énergétique ouvre le bénéfice du taux de 5,5 %, les autres travaux étant taxés à 10 %. L'Union sociale pour l'habitat (USH) estime que moins de 50 % des travaux d'économies d'énergie réalisés par les bailleurs sociaux bénéficient du taux de 5,5 %. %. L'objectif de notre amendement est d'élargir l'application de ce taux à l'ensemble des travaux d'économies d'énergie, comme cela a été le cas entre 2014 et 2018. La parole est à M. Pascal Savoldelli,

M. Rémi Féraud. Cet amendement vise à faire passer de 20 % à 10 % le taux de TVA pour les travaux de surélévation d'un immeuble existant.

est à Mme Valérie Létard. La crise sanitaire a mis en exergue l'urgente nécessité de loger à proximité de leur lieu de travail, et moyennant des loyers abordables, les agents ou salariés du secteur public qui contribuent de manière essentielle à la continuité des services publics, notamment les personnels soignants, les postiers ou les agents d'EDF. Le logement intermédiaire répond à ce besoin économique et social majeur, en proposant des loyers entre 10 % et 15 % inférieurs aux prix du marché. Il constitue une offre de logements adaptée à ces personnes clés, issues des classes moyennes, qui connaissent des difficultés croissantes d'accès au logement à proximité de leur lieu de travail, en particulier dans les zones tendues. Par conséquent, et pour favoriser la production de logements intermédiaires, il est proposé de modifier l'article 279-0 A du code général des impôts pour faire bénéficier du régime fiscal du logement intermédiaire les opérations portant sur des logements loués à l'État, à ses établissements publics ou à des entreprises publiques, telles que La Poste ou EDF, dès lors que ces logements sont destinés à être occupés par ceux de leurs agents ou salariés qui sont éligibles au logement intermédiaire. En l'état actuel de la législation, les logements intermédiaires doivent être loués à des personnes physiques sous conditions de revenus

Il s'applique, de manière générale, à des logements destinés à des personnes dont les ressources n'excèdent pas certains plafonds, supérieurs à ceux du logement social. Ces personnes doivent être locataires du logement visé. visé. Votre amendement vise le cas où des personnes respectant ces conditions ne sont pas directement locataires, mais occupent un logement loué par l'État, l'un de ses établissements publics ou une entreprise publique.

la réussite de ce programme : à l'heure où les villes moyennes connaissent un regain d'attractivité auprès des populations, en particulier des classes moyennes, qui aspirent à une autre qualité de vie, ce programme a montré son intérêt.

c'est-à-dire aux communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d'ORT. Il ne s'agit pas d'une mince

Mme Isabelle Briquet. Le mécanisme du bail réel solidaire (BRS), créé en 2016, vise à favoriser des opérations d'accession sociale, en instituant une dissociation de la propriété du foncier et du bâti et en garantissant une quasi-pérennité de l'affectation du logement à la résidence principale des ménages à revenus modestes. Compte tenu de ces caractéristiques, le législateur a prévu que les opérations de BRS bénéficient du taux réduit de TVA de 5,5 Parallèlement, l'article 284 du code général des impôts prévoit que, si les conditions d'application du taux réduit cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent l'acquisition des droits par le ménage, l'organisme de foncier solidaire devra reverser au Trésor public le différentiel de TVA. L'organisme de foncier solidaire est donc garant du maintien de l'affectation du logement et du respect, par les ménages acquéreurs, des règles encadrant ce dispositif. Cela étant, si le manquement à ces règles est imputable au ménage, il convient de ne pas sanctionner l'organisme de foncier solidaire avant de lui avoir laissé le temps de régulariser la situation. Les dispositions du code de la construction et de l'habitation lui permettent, en cas de manquement de ce type, d'obtenir la résiliation du bail réel solidaire et de signer ensuite un autre BRS avec un nouveau ménage sous plafond de ressources. Il est proposé de laisser à l'organisme de foncier solidaire un délai maximum de deux ans pour effectuer cette régularisation avant d'appliquer la sanction.

L'article 9 de ce projet de loi propose la prorogation jusqu'au 31 décembre 2022 du relèvement du seuil de chiffre d'affaires en deçà duquel les assujettis à la TVA installés en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion bénéficient du dispositif de franchise en base de TVA.

Si l'objectif de cet article est louable, rien dans l'exposé des motifs ou la discussion de l'amendement à l'Assemblée nationale ne justifie le choix de prolonger de seulement huit mois ce dispositif.

Je ne suis pas toujours très favorable à ce type de dérogation, mais il s'agit de permettre à nos compatriotes qui partent vivre dans un pays

n° I-133 rectifié. Cet amendement a pour objectif d'exonérer d'impôt sur les sociétés et de contribution économique territoriale l'activité en bail réel solidaire des organismes de foncier solidaire (OFS). Ces organismes sont sans but lucratif, agréés et contrôlés par le représentant de l'État en région, aussi bien sur le respect de la réglementation propre à leur activité que sur les principes spécifiques de gestion, définis par un décret en conseil d'État, qui leur imposent notamment de prévoir dans leurs statuts un réinvestissement intégral de leurs bénéfices dans leur activité de BRS. À ce titre,

Or leur régime d'imposition à l'impôt sur les sociétés ou à la contribution économique territoriale peut varier en fonction de la forme choisie, certains étant exonérés, d'autres non. Compte tenu de leur mission d'intérêt général et afin d'harmoniser leur régime, il est proposé de prévoir, au profit de tout organisme de foncier solidaire, une exonération d'impôt sur les sociétés et une exonération de contribution économique territoriale.

n° I-133 rectifié. Cet amendement a pour objectif d'exonérer d'impôt sur les sociétés et de contribution économique territoriale l'activité en bail réel solidaire des constitués sous forme de société coopérative d'intérêt collectif. Sur un plan juridique, ces organismes peuvent être constitués sous diverses formes.

ne fasse pas obstacle à ce que ces sociétés puissent accéder aux mêmes avantages que les associations, notamment en matière fiscale.

soit à d'autres cessionnaires qui s'engagent à réaliser des logements sociaux dans les quatre ans. Les organismes de foncier solidaire peuvent bénéficier de ce régime, mais sont actuellement soumis au délai de quatre ans, et non à celui de dix ans prévu pour les organismes de logement social. Or ils sont amenés, comme les organismes HLM, à intervenir dans des opérations complexes qui peuvent nécessiter un délai supérieur à quatre ans. Le dispositif des baux réels solidaires est devenu l'outil antispéculatif des collectivités qui veulent agir au service de l'accession à la propriété des ménages à revenus modestes. Il a vocation à se développer sur tous les territoires, dès lors qu'il existe un enjeu de maîtrise du foncier. Nous devons donc faire en sorte d'accompagner

En dehors de ces cas, les organismes de foncier solidaire concourant à la conclusion d'un bail réel bénéficient d'une exonération suivant le régime applicable à tout autre cessionnaire.

n° I-96 rectifié. Afin de soutenir la création de logements sociaux, le code général des impôts prévoit une exonération d'impôt sur les plus-values en faveur des personnes physiques lors des cessions d'immeubles, lorsque l'acquéreur s'engage ensuite à réaliser des logements sociaux.

effet conduit à exclure du dispositif des opérations d'acquisition-amélioration réalisées par les bailleurs sociaux, qui y étaient éligibles auparavant.

est l'avis du Gouvernement ? L'inclusion des opérations de rénovation-amélioration dans le champ des exonérations ne serait pas en adéquation avec l'objectif du dispositif, qui est de favoriser les opérations immobilières d'ampleur se traduisant par la production de nouveaux logements sociaux.

Cette situation encourage la spéculation immobilière et pousse certains propriétaires à conserver leurs locaux vacants dans l'attente de plus-values toujours plus importantes. Pour les entreprises, la possession de locaux vacants est même parfois un élément apprécié par les investisseurs

et que la France vient d'accueillir le Congrès mondial de la nature de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), l'article 10 du projet de loi de finances pour 2022 prévoit la suppression de la réduction d'impôt sur le revenu pour dépenses d'entretien des espaces naturels protégés. Dans les faits, on assiste à la disparition d'une incitation à gérer, entretenir et restaurer les aires protégées et à une nouvelle hausse de la taxation des aires protégées, après celle de 2018. Selon une technique classique, ce régime fiscal avait été progressivement rogné dans plusieurs projets de loi de finances successifs, jusqu'à le rendre squelettique et donc peu attractif. Il est ainsi plus facile pour le Gouvernement de le déclarer improductif. La bonne réforme serait, au contraire, de le rendre efficace ! C'est pourquoi cet amendement tend à revenir sur la suppression de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées sur certains espaces naturels en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel. Si le Gouvernement veut se montrer cohérent avec ses orientations sur l'augmentation des surfaces protégées, nous l'invitons à rehausser le niveau d'attractivité de cette disposition fiscale, afin qu'elle ne soit plus sous-employée par les contribuables.

tout, en partie ou « en mélange » des habitats naturels. Ces habitats sont ceux pouvant faire l'objet d'interdictions de destruction, de coupe, de prélèvement, de cueillette, d'altération ou de dégradation, ainsi que de toute autre pratique ayant un impact sur eux au titre des directives Oiseaux et Habitats. Ce sont également les habitats susceptibles de faire l'objet d'arrêtés de protection de biotope et, plus largement, d'arrêtés portant protection des habitats naturels. Contrairement aux forêts, ces milieux sont essentiellement non productifs et ne génèrent pas de revenus pour leurs propriétaires.

des taux communautaires de taxe d'habitation sur une période pouvant aller jusqu'à douze ans. Cette possibilité a permis de limiter l'augmentation de la pression fiscale subie par les contribuables des communes entrantes, lorsque les taux d'imposition additionnels étaient largement supérieurs aux taux des communes rattachées, ne permettant pas une baisse des taux communaux correspondant au transfert de charges. L'article 29 de la loi de finances pour 2021 a prévu les modalités de réduction de la taxe sur le foncier bâti (FB) et de la cotisation foncière des entreprises des établissements industriels évalués selon l'article 1499 du code général des impôts. Le calcul de la compensation perçue par les EPCI à fiscalité propre est réalisé à partir des taux de foncier bâti et de CFE appliqués sur le territoire en 2020. En retenant le taux appliqué en 2020, l'article 29 induit une moindre compensation pérenne de la diminution des impôts de production pour les EPCI ayant dû recourir au dispositif de lissage des taux pour permettre la mise en oeuvre des nouvelles cartes intercommunales. Afin de limiter cette perte de recettes pour les EPCI concernés, il est proposé d'intégrer, pour le calcul de la compensation, les fractions annuelles de taux appliquées sur le territoire des communes concernées jusqu'au terme de la période d'harmonisation, sans retenir les éventuelles décisions d'augmentation des taux de l'EPCI. Ainsi, à l'issue de la période d'harmonisation, le taux retenu correspond au taux qui aurait été appliqué sur le territoire de l'EPCI en 2020 en l'absence de processus d'harmonisation.

Dans ce cas, quand une commune a rejoint un EPCI, le code général des impôts permet d'instituer un mécanisme de rattrapage progressif de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Pourtant, les taux pris en compte dans le cadre des réformes des impôts de production sont les taux observés en 2020, ce qui induit une forme de sous-compensation pérenne par rapport au produit que la commune aurait pu percevoir une fois la trajectoire atteinte. Pour autant, cette perte de ressources me paraît assez virtuelle, puisque, finalement, elle survient au terme d'une trajectoire qui n'a pas été imposée à l'EPCI. Ce cas ne me paraît donc ni constituer

cet amendement qui visait à supprimer deux petites taxes inutiles. Il y a des années, lorsque le TGV était en plein essor, il a été décidé de taxer la SNCF

alors que notre groupe avait demandé, dans cet hémicycle, que ce soit le taux de 2020 qui soit retenu. Ce paramètre était particulièrement important, car il était prévu un mécanisme de remise à charge pour les communes et intercommunalités ayant augmenté leur taux de taxe d'habitation entre 2017 et 2019.

de règlements départementaux ayant de lourdes conséquences financières pour un certain nombre de communes rurales. La mobilisation de la totalité du budget d'investissement sur toute la mandature est parfois nécessaire, comme nombre de maires ont pu le signaler au président du Sénat lors de ses déplacements.

ils estiment qu'une habitation sur trois en zone rurale n'est pas couverte en défense incendie, et ils évaluent à 1,2 milliard d'euros sur trois ans le besoin de financement induit par la mise aux normes pesant sur les communes. Le rapport préconise d'abonder en conséquence le plan de relance d'une première tranche de 400 millions d'euros pour aider les communes à financer ces travaux, la mise aux normes défense incendie ayant également comme vertu de débloquer un certain nombre de projets de construction dans nos territoires et d'être ainsi bénéfique à la relance économique de notre pays. Toutefois, compte tenu de l'absence

à l'instant vise à ajouter un nouveau cas de dérogation pour les communes qui ont augmenté leur taux de taxe d'habitation pour financer l'exercice de nouvelles compétences suite d'un changement d'EPCI, dès lors que le total des produits communaux et intercommunaux prélevés sur le territoire de la commune n'a pas varié. L'idée est pertinente, et son esprit est conforme à celui de l'article 10 , puisque la condition d'un non-accroissement de la pression fiscale

nous estimons que la référence au taux de l'année 2017 permet, dans la lignée des dispositions de la loi de finances initiale pour 2018, à la fois de garantir le maintien des ressources des collectivités territoriales et d'atténuer le coût pour les finances publiques de la réforme de la taxe d'habitation. Adopter cet amendement ouvrirait une brèche dans l'équilibre financier général de la compensation. Quel est maintenant l'avis

a étudié et confirmé dans un rapport publié en juin 2019 le caractère excessif de la taxation appliquée aux titres de séjour. Ainsi, la France applique la deuxième taxation la plus élevée en Europe pour les titres de séjour délivrés aux résidents de longue durée.

des dispositions relatives aux collectivités territoriales- communes, intercommunalités, départements et régions -et fixe pour 2022 la dotation globale de fonctionnement (DGF), ainsi que les variables d'ajustement.

et une minoration des variables d'ajustement difficilement justifiable dans le contexte actuel. Néanmoins, nous soutiendrons cet article. Mes

la dotation globale de fonctionnement afin de permettre aux collectivités territoriales, en particulier aux communes rurales, de se doter de moyens supplémentaires en ingénierie. Ces moyens sont indispensables, par exemple, pour le déploiement et l'animation territoriale des ou pour mener les investissements prévus dans le cadre du plan de relance. Nous le savons, nombreuses sont les collectivités territoriales qui connaissent une carence en ingénierie de projet, et ce en dépit des besoins accrus qui se font sentir sur les territoires. L'amendement n° I-520,

Madame la ministre,

aux AOM. Le maintien d'un tel plafonnement est difficilement compréhensible, alors même que les AOM enregistrent des pertes financières importantes en raison de la crise sanitaire et que la compensation avait atteint 91 millions d'euros en 2019. Il est nécessaire de garantir un dispositif de soutien financier équitable entre les autorités organisatrices de la mobilité, quelles que soient leur forme juridique et leur localisation géographique, même loin de la capitale.

l'heure. Voilà cinq ans, ces variables d'ajustement s'élevaient non pas à 50 millions d'euros, mais à 870 millions, et elles touchaient toutes les strates de collectivités locales. Comme les régions, les AOM n'ont jamais été oubliées.

Ces opérations représentent généralement des montants d'investissement élevés. Ainsi, leur non-éligibilité au FCTVA entraîne mécaniquement une perte de recettes importante, qui va réduire la capacité des collectivités à financer leurs projets d'investissement, fait leur participation à la relance économique. En outre, nombre de ces opérations correspondent à des enjeux de transition écologique. Accompagner ces opérations en les réintégrant dans le champ du FCTVA apparaît donc pleinement cohérent

Pour être pleinement efficace, cette mesure ne devra pas être neutralisée par l'exclusion d'autres dépenses du champ du FCTVA.

La définition du périmètre des dépenses automatisées a conduit à rendre certains comptes de classe 2 inéligibles

Ces dépenses peuvent représenter un coût important pour les collectivités, en particulier en milieu rural et en zone de montagne, où l'offre de prestataires est souvent faible, ce qui empêche une négociation des tarifs. Dans une réponse à une question écrite du 4 avril 2019, la ministre de la cohésion des territoires avait indiqué que les dépenses de déneigement constituaient des dépenses de fonctionnement en vertu d'une circulaire du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local.

à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Ce texte prévoit un montant plafond, mais aucun montant plancher,

Cet amendement vise à inclure dans ce mécanisme les pertes de recettes tarifaires subies par les communes rurales, consécutives à la non-exploitation des salles communales pendant la crise sanitaire.

aux communes de moins de 1 000 habitants, dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,25 fois le potentiel des communes de la même strate, et aux salles communales de ces communes construites depuis cinq ans au plus

du 19 juillet 2021. À ce titre, deux dotations ont été créées : une dotation de compensation des pertes d'épargne brute subies par les régies et une dotation de compensation des pertes de recettes tarifaires.

Malgré cela, l'État n'a pas augmenté sa contribution financière. La charge nette pour les départements a donc accusé une hausse globale de 15 %. L'ODAS estime que « l'accroissement du nombre d'entreprises en difficulté amènera fin 2021, et surtout en 2022, un afflux de nouvelles demandes de RSA

un reste à charge total de 4,6 milliards d'euros. Les départements assument les conséquences, non seulement de la conjoncture, mais aussi des mesures prises nationalement. Par exemple, lorsque l'État a décidé unilatéralement d'attribuer le RSA aux salariés suspendus, car non vaccinés, ce sont bien les départements qui ont dû soudainement en assumer le coût.

entendons prendre en compte la situation des départements qui, en 2022, verront leurs dépenses d'allocation du RSA augmenter de plus de 5 % par rapport à

Pour résumer, en 2022, les collectivités territoriales percevront de l'État la CVAE acquittée en 2021 par les entreprises, mais pour le solde de l'année 2020. Dans ses dernières actualisations, le député Jean-René Cazeneuve, chargé de suivre les effets de la crise sur les finances locales, estime que la baisse de la CVAE,

de nombreux ménages. Il s'agit donc d'une mesure de justice sociale qui répond parfaitement à l'urgence de la crise sanitaire. Il est logique que les plus aisés participent à l'effort pour l'intérêt général.

près qu'il concerne la taxe d'habitation communautaire. L'article 16 de la loi de finances pour 2020 a prévu les modalités de suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales et l'introduction d'un nouveau schéma de financement des collectivités locales à compter de 2021. Le calcul de la compensation perçue par les EPCI à fiscalité propre est réalisé à partir du taux de taxe d'habitation intercommunal appliqué sur le territoire en 2017 et de la base d'imposition 2020 des locaux meublés affectés à l'habitation principale. En retenant le taux appliqué en 2017, l'article 16 ne tient pas compte de la mise en oeuvre progressive du taux de taxe d'habitation sur le territoire des communes rattachées et induit une moindre compensation pérenne de la réforme fiscale. Afin de limiter cette perte de recettes pour les EPCI concernés, et compte tenu de l'interruption des lissages de taux de taxe d'habitation à partir de 2020, nous proposons d'intégrer au calcul les fractions de taux des années 2017 à 2019 appliquées sur le territoire des communes concernées, sans retenir les éventuelles décisions d'augmentation du taux de l'EPCI. Quel est l'avis de la commission

à fiscalité propre correspond à la somme de « la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020

et institue un nouveau schéma de financement des collectivités locales. Cette réforme a des conséquences sur le financement des syndicats de communes et, par ricochet, sur la situation des contribuables locaux. En effet, plusieurs communes membres de ces établissements publics ont choisi de recourir à une fiscalisation des contributions devant être versées aux syndicats de communes. Dans ce cadre, le montant de la contribution versée au syndicat est recouvré comme une taxe additionnelle à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la La suppression de la taxe d'habitation est donc susceptible d'entraîner un ressaut d'imposition au détriment des contribuables fonciers. Cet amendement vise à neutraliser les conséquences de la réforme pour les contribuables concernés

tend à minorer chaque année le montant des contributions à recouvrer sur le territoire des communes concernées de la part correspondant à la taxe d'habitation sur les résidences principales en 2020, afin d'éviter le ressaut d'imposition des contribuables fonciers. Quel est l'avis de la commission

Cela peut constituer une solution pour les départements qui le demandent. En revanche, notre groupe exprime le souhait que soient recentralisés non pas le seul financement du RSA, qui est le coeur du problème, mais aussi l'instruction des dossiers et la décision d'attribution. Nous craignons en effet que le département, qui est chef de file de l'action sociale, notamment dans la lutte contre le non-recours aux prestations sociales, n'y perde une partie de son identité. Nous craignons également que la proximité permise aujourd'hui par son action ne disparaisse progressivement

Certes, le département de Seine-Saint-Denis retrouvera une épargne brute. Mais elle aurait été beaucoup plus importante si nous étions dix ans plus tôt et s'il n'y avait pas eu ces conditions de décentralisation.

y a une proposition d'expérimentation avec un accord passé entre le Gouvernement et le département. Je me suis personnellement assuré

propose aux départements et aux collectivités exerçant la compétence d'expérimenter le transfert à l'État de l'instruction administrative, de la décision d'attribution et du financement du RSA. Cette expérimentation doit concourir au renforcement des politiques d'insertion des collectivités qui s'engageraient dans cette voie. le dispositif issu de la discussion à l'Assemblée nationale pose deux difficultés importantes. D'une part, il est prévu, à titre de compensation de la recentralisation du RSA, qu'un certain nombre de ressources puissent être retenues, donc non versées. D'autre part, le Gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale, à l'occasion de l'examen de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », un amendement qui vise à neutraliser les effets d'une recentralisation de l'allocation de RSA. Concrètement, une partie du coût de la recentralisation

Au contraire, elle en menace le fonctionnement et l'adhésion de l'ensemble des départements à la péréquation horizontale interdépartementale.

examiner la situation de la défense incendie, spécifiquement dans les communes rurales. Ils ont conclu qu'il convenait d'investir rapidement, sous trois ans, 1,2 milliard d'euros pour

que de très nombreux urbains et métropolitains quittent les grandes villes pour s'installer et travailler dans des territoires ruraux, le fait qu'ils ne puissent pas le faire au motif que les communes ne peuvent parfois pas leur délivrer des permis de construire est un véritable problème.

de flécher la dotation vers des dépenses spécifiques, alors que son attribution est confiée aux préfets, dans le respect des priorités fixées par la commission des élus pour la DETR.

notamment la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints, les autorisations d'absence et les frais de formation des élus. En métropole, la dotation est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants sous condition de potentiel financier avec un plafond actuellement fixé à 1,25 fois le potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants. En raison de la condition liée au potentiel financier, près de 3 000 communes ne perçoivent pas la dotation. En effet, le potentiel financier d'une commune est calculé en intégrant fictivement une partie des ressources de son EPCI. EPCI. Cet amendement vise donc à supprimer la condition de potentiel financier pour les communes de moins de 1 000 habitants.

Cette subvention est répartie par l'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif et après avis du représentant de l'État, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen d'un rapport annuel établi par le président du conseil exécutif. » En Corse, les crédits relatifs à la montagne font donc l'objet, dans des conditions déterminées en loi des finances, d'une subvention globale à la collectivité territoriale de Corse.

Pourriez-vous par ailleurs nous répondre sur la prépondérance que le représentant de l'État s'est octroyée en outrepassant son rôle administratif en se prononçant sur la répartition de ces dotations par l'assemblée de Corse en tant que commissaire de massif, ce à contresens de l'esprit des textes ? Pour précision, il n'y a pas de commissariat de massif en Corse, car c'est l'administration de la collectivité de Corse qui fixe les règles de fonctionnement et la composition du comité de massif. le représentant de l'État agit de la sorte, y compris en freinant les projets ou en prenant à son compte en tant que prétendu commissaire du massif le plan montagne, en cours de déploiement, comme tout plan de relance.

Cet amendement vise à relever le financement de la dotation de continuité territoriale à plusieurs titres : aider les compagnies délégataires à faire face à la crise du covid-19, leur permettre de poursuivre la politique de baisse tarifaire initiée pour le fret

Sur ce dernier point, je me fais ici le relais du vote qui a eu lieu vendredi dernier à l'assemblée de Corse. Celle-ci n'a pas inscrit au budget supplémentaire la somme de 86 millions d'euros qu'elle a été condamnée à payer. Avant d'aborder la question du droit et du budget, une question fondamentale qui doit être posée : celle de la responsabilité et de la morale en politique.

C'est donc l'État lui-même qui a été tout à la fois chef d'orchestre et bénéficiaire de ce détournement. Il s'agit là d'une responsabilité historique. Le vote qui a eu lieu à l'assemblée n'est pas celui d'une Corse qui s'oppose ou refuse le dialogue. C'est celui d'une Corse qui refuse le poids et le fardeau de l'injustice, le poids d'une privation organisée par l'État et dont les Corses paient les conséquences quinze années plus tard. Inscrire ces 86 millions d'euros, c'est reconnaître la responsabilité totale et entière de la collectivité et faire peser sur les Corses le poids d'un mensonge et d'une injustice : celle de responsabilités qui ne lui reviennent pas.

Monsieur Parigi, votre amendement me paraît poser une difficulté d'ordre juridique, puisque la dotation de continuité territoriale de Corse est une mesure budgétaire, et non un prélèvement sur recettes.

Même avis, pour les mêmes raisons. Monsieur Parigi, j'ai porté attention aux débats que j'ai pu avoir avec les députés de Corse à l'Assemblée nationale. Le travail continuera avec eux, ainsi qu'avec l'ensemble des élus.

des ressources (FNGIR), qui a été mis en place pour neutraliser la réforme fiscale ayant accompagné la suppression de la taxe professionnelle, notamment le transfert de la taxe d'habitation des départements vers le bloc communal.

Mme Isabelle Briquet. Cet amendement vise à supprimer les économies faites sur les divers organismes chargés de missions de service public ponctionnés par le présent projet de loi de finances 37 millions d'euros sur la dotation de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France ; 45 millions d'euros sur la dotation du Fonds national d'aide au logement 30 millions d'euros sur la dotation de l'Institut national de la propriété industrielle ; 200 000 euros sur la dotation de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ; et un total de 22 millions d'euros sur les dotations de plusieurs établissements publics fonciers régionaux. Notre groupe s'oppose au démantèlement de la puissance publique engagée par le Gouvernement, qui fragilise depuis 2017 les administrations centrales et leurs opérateurs.

sur l'initiative de Ronan Dantec, vise à rehausser le plafond mordant pour les agences de l'eau à un niveau correspondant aux moyens annuels dont elles disposaient pour la période 2013-2018. Il s'agit d'éviter le report ou la suppression de dispositifs d'aides qui sont nécessaires à la bonne gestion de l'eau dans les territoires.

en matière de protection de la ressource. Les auteurs de ce rapport constatent que le plafond mordant et sa dynamique sont à l'origine d'une baisse structurelle des moyens des agences de l'eau. Or les collectivités ont besoin de l'aide des agences de l'eau, car il reste beaucoup à faire, notamment en raison du risque climatique.

étendu, notamment à la lutte contre le changement climatique. Cet amendement vise à rehausser le plafond mordant à 2 351 000 euros, au lieu de 2 197 620 euros, ce qui permettrait de remédier à la baisse de capacité d'action des agences de l'eau.

Cozic. Cet amendement vise à allouer 844,56 millions d'euros des recettes de la taxe sur les transactions financières (TTF) à l'aide publique au développement. Cette somme correspond à 51 % des recettes totales prévues pour la TTF pour l'année 2022, soit 1,656 milliard milliard d'euros. Je rappelle les engagements du Gouvernement, traduits à l'alinéa 10 de l'article 1 de la loi du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Dans un souci de conciliation, le Sénat a dû renoncer à sa volonté de porter à 51 % la part du produit de la taxe sur les transactions financières à destination du fonds de solidarité et de développement (FSD) en échange d'un maintien du produit de la TTF à un montant qui ne peut pas être inférieur à 528 millions d'euros

clair : assécher financièrement l'audiovisuel public par le biais des dotations, mais aussi de la fiscalité affectée. La désindexation de la contribution, qui n'apporte aucun gain de pouvoir d'achat pour les ménages, a un coût réel pour les opérateurs estimé à plus de 50 millions d'euros.

libéralisant un peu plus les opérateurs. Pour la baisse des dotations et des ressources fiscales, le compte est bon, si l'on peut dire : depuis 2018, ce sont près de 200 millions d'euros de dotations qui ont disparu, auxquels il faut ajouter les dégrèvements de la redevance télé, estimés à 625 millions d'euros, soit la diminution de ladite redevance de 1 euro et les deux années de désindexation. Mais du côté des nouvelles ressources, l'abandon du grand projet de loi sur l'audiovisuel public a fortement limité leur impact. Le seul atout marquant, négocié à l'échelon européen, sera donc la contribution des plateformes à la production. Pourtant, il faut rappeler deux choses essentielles. Premièrement, et c'est d'ailleurs un point saillant du rapport de nos collègues députés, la redevance française fait partie des plus faibles d'Europe. Deuxièmement, il apparaît d'autant plus nécessaire, dans ce contexte de montée des discours dangereux, de donner une réelle assise à un service public audiovisuel.

mais de réussir à fidéliser ceux qui sont déjà abonnés. La conjoncture économique laisse craindre une baisse non négligeable du pouvoir d'achat. Le risque, dans ce contexte, est de voir certains abonnements annulés, considérés comme des dépenses annexes. Il y a donc un intérêt pour les publications à ce que la souscription d'abonnements soit facilitée.

théorie, les professions libérales peuvent bénéficier de cette déduction. Cependant, les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux (BNC) n'ont pas la faculté de créer au passif de leurs bilans un compte de réserve et ne peuvent ainsi pas satisfaire

dans le cadre de la détermination du résultat fiscal. Sont entre autres concernés les avocats, les notaires, les médecins, les dentistes et les professions paramédicales. Or ces professionnels reçoivent des personnes privées à titre régulier et ils sont nombreux à vouloir soutenir les artistes en achetant leurs oeuvres et en exposant celles-ci, diffusant par là le travail de leur art.